J'aimerais à mon tour exprimer toute notre reconnaissance envers les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces engagées, notamment les élus locaux, pour lutter contre les flammes. La Gironde n'est malheureusement pas la seule touchée. Partout en France et en Europe, les feux ravagent les territoires, dans un contexte marqué par des chaleurs très fortes et d'importantes sécheresses. Avec le réchauffement climatique, le risque d'incendie devrait s'intensifier et s'étendre plus largement sur le territoire national au cours des années à venir. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques ont opportunément créé, voilà trois mois, une mission d'information sur ce sujet, contribue, sera très prochainement publié. Il contiendra un certain nombre de propositions fortes pour intensifier, en urgence, la lutte contre les feux extrêmes et mieux les prévenir. Cela passe par le renforcement de notre flotte aérienne, l'adaptation à la remontée vers le nord du risque d'incendie, la garantie du recrutement et de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, l'indispensable participation financière de l'État aux investissements des l'engagement d'une réflexion transversale en matière de prévention, la poursuite des efforts relatifs aux obligations légales de débroussaillement, l'adaptation de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire face à l'aléa, une gestion forestière adaptée au risque et le renforcement massif de la sensibilisation des Français à cette question. Madame la ministre, l'heure est très grave ; j'en appelle à la mobilisation générale Le Gouvernement est-il prêt, d'une part, à étudier sans délai ces axes de réflexion, dans le cadre d'une stratégie interministérielle abordant l'ensemble des pistes en matière tant de prévention que de lutte,

d'une extrême difficulté, parfois au péril de leur vie, pour protéger les populations et les territoires de l'avancée du feu. Monsieur le sénateur, vos questions se rapportent à notre modèle de sécurité civile, dont vous êtes, je le sais, un parfait connaisseur. La solidarité nationale que vous appelez de vos voeux est déjà à l'oeuvre. Ainsi, en Gironde, les renforts nationaux représentent actuellement plus de 1 200 personnes, trois détachements à pied, colonnes « feux de forêt », deux groupes urbains, une colonne lourde « feux de forêt » et un groupe d'appui tactique. Cette solidarité nationale est essentielle dans une telle crise. moi aussi, saluer le rôle des élus locaux, que j'ai eus, personnellement et individuellement, au téléphone, hier et avant-hier. Leur rôle est essentiel et je tiens à les remercier. Départements et communes sont en effet des acteurs majeurs de notre modèle de sécurité civile et de lutte contre les incendies. Monsieur le sénateur, les réflexions que vous conduisez seront utiles pour penser les lendemains de cette crise avec l'ensemble des acteurs. de nouveau de la mobilisation du Gouvernement, avec l'ensemble des forces impliquées dans cette crise. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la sécheresse que nous subissons est le combustible idéal pour les feux de forêt. Après l'incendie de la Montagnette, dans les Bouches-du-Rhône, et celui des monts d'Arrée- du jamais vu ! -, dans le Finistère, c'est aujourd'hui, malheureusement, la Gironde qui brûle. Les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, sapeurs ou marins, et que je tiens à saluer ici, font face à ces feux avec un grand courage. J'ai aussi une pensée pour les populations, qui, pour certaines, ont perdu beaucoup dans les flammes. L'engagement des communistes que nous sommes en la matière n'est pas nouveau. En prenant la parole aujourd'hui, je m'inscris dans la continuité du travail réalisé, en son temps, par mon prédécesseur Louis Minetti, qui avait d'ailleurs abouti à une loi portant son nom en 1991.

outre la sécheresse estivale et le réchauffement climatique, l'une des principales causes des feux est l'absence de gestion durable des forêts. Le pastoralisme était autrefois un moyen efficace pour nettoyer les bois et réduire les risques de départ de feu. Pour chaque région, des réflexions concertées avec l'ensemble des acteurs concernés doivent être engagées pour trouver des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire. Des régions qui n'étaient pas menacées auparavant sont aujourd'hui affectées par la sécheresse. Hier encore, nous pouvions déplacer des moyens humains et matériels d'un département à l'autre. Aujourd'hui, cela n'est plus possible, tant le risque d'incendie est grand, y compris dans des départements jusque-là épargnés par les flammes. Madame la secrétaire d'État, la quantité de Canadair et d'autres engins de lutte doit-elle rester la même aujourd'hui qu'hier ? Les 5 000 pompiers non vaccinés, suspendus de leurs fonctions, ne manquent-ils pas pour lutter contre les incendies ? Face à ces nouvelles réalités, puisque nous sommes en guerre contre le feu, seriez-vous disposée à créer une véritable cellule de crise transpartisane visant à mettre en place un plan de lutte adéquat, associant l'ensemble des acteurs, notamment la filière bois et les communes, et tenant compte des spécificités de chaque territoire ? La parole

le Président de la République sera à leurs côtés dès cet après-midi. À chaque incendie, c'est tout un écosystème forestier qui est dévasté, toute une biodiversité qui est menacée et tout un puits de carbone qui est anéanti.

et nous devons intensifier les outils et moyens mis en oeuvre dans les régions du Sud et les étendre à l'ensemble du territoire. Je pense aux 200 plans de prévention des risques d'incendie de forêt, mais également à la politique de défense de la forêt contre les incendies du ministère de l'agriculture. Dans cette perspective, les obligations légales de débroussaillement sont un maillon essentiel, mais elles ne se sont pas appliquées partout comme elles le devraient ; on le constate notamment avec le feu de La Teste-de-Buch, en Gironde.

Par ailleurs, si le changement climatique accroît les risques d'incendie, je dois rappeler que 90 % des incendies sont d'origine humaine, que ce soit par imprudence ou par malveillance.

comme chaque année, l'attente des jeunes et de leur famille vis-à-vis de Parcoursup est grande et peut susciter une forme d'inquiétude. En effet, cette plateforme permet aux bacheliers de décider de leur avenir dans les études supérieures. Les lycéens sont invités à formuler jusqu'à trente voeux, sans les classer. Une commission d'examen est ensuite désignée dans chaque unité de formation et de recherche. Il n'y a pas, pour le moment, d'algorithme unique de sélection ; en 2020, la Cour des comptes proposait de rendre publics les algorithmes locaux. Les lycéens sont ensuite invités à accepter ou à décliner chaque offre, sous quatre jours, ce qui libère des places pour d'autres. Ils doivent donc rester vigilants tout au long de la procédure. Depuis le jeudi 2 juin, les lycéens ont reçu leurs premières réponses. Le 23 juin, ils ont pu formuler jusqu'à dix nouveaux voeux. Certains ont attendu jusqu'au 15 juillet pour connaître leur affectation. Aux dernières nouvelles, 86 % des élèves de terminale et 71,6 % des étudiants en réorientation ont reçu une réponse. C'est bien mieux qu'en 2021.

Madame la ministre, le processus de Parcoursup s'est terminé voilà quelques jours. Pouvez-vous nous présenter le bilan que vous en avez fait, nous indiquer comment les rectorats vont accompagner les candidats qui n'ont pas encore eu de proposition et nous présenter les améliorations que vous envisagez d'apporter pour l'an prochain ? La parole

La parole est à M. Hervé Gillé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Aucune victime n'est à déplorer dans ce contexte, c'est remarquable ! Je remercie également le président du Sénat de sa visite et du temps nécessaire qu'il a consacré à écouter l'ensemble des acteurs, plus particulièrement les élus locaux.

propriétés de l'État, a été déléguée à un prestataire privé. Seulement quatre avions Dash sur six et neuf Canadair sur douze sont en mesure de voler ; les deux tiers ont plus de 25 ans. Nous luttons contre la crise climatique avec des moyens du siècle passé la secrétaire d'État, comptez-vous renforcer la flotte européenne et nationale et relocaliser au moins deux Canadair dans le Sud-Ouest ? Comptez-vous contribuer à la création d'un secrétariat d'État aux risques civils et crises majeures ?

Oui, monsieur le sénateur Gillé, nous vivons tous actuellement au rythme des incendies qui ravagent notre territoire et je vous sais particulièrement sensible à ceux qui touchent le département Permettez-moi d'abord de m'associer à l'hommage que vous et d'autres orateurs avez rendu à nos pompiers investis, mais également- il ne faut pas les oublier -aux militaires, aux élus, aux gendarmes et aux policiers très largement mobilisés sur ces feux de forêt depuis le 12 juillet dernier. Chacun se sent concerné par ces événements.

La difficulté, nul ne l'ignore, réside dans le feu, particulièrement important, qui sévit en Gironde- c'est d'ailleurs l'objet de votre question, monsieur le sénateur. Le dernier grand incendie que nous avons connu en Gironde a touché 700 hectares

qui vous interrogeait pertinemment sur la colère provoquée par la rédaction des décrets d'application de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), vous avez évoqué « un manque d'accompagnement et de pédagogie vis-à-vis des élus locaux Au-delà de la formule, quelque peu paternaliste à l'endroit des maires et de leurs conseillers municipaux, nous ne vous tiendrions pas rigueur de ce « manque » si l'enjeu n'était pas de taille. En effet, il y va de l'avenir de nos territoires et en particulier de la ruralité, qui souffre d'un manque d'attractivité en raison de l'impossibilité pour certaines communes de proposer des terrains constructibles à de nouveaux arrivants. Cette réalité est d'autant plus frustrante que nous percevons le retour en grâce de la vie en milieu rural depuis la crise sanitaire.

autre incertitude m'a été signalée par quelques intercommunalités du département dont je suis élue, la Lozère, qui, malgré des efforts considérables de partage, de coconstruction, de plans d'aménagement et de marketing territorial, passeront bientôt sous le seuil fatidique des 5 000 habitants, ce qui mettra en péril leur périmètre et, partant, leur existence.

Une telle augmentation à l'échelon mondial signifie une hausse des températures d'environ 4 degrés en France, soit plus du double du réchauffement aujourd'hui constaté dans notre pays, qui se situe autour de 1,8 degré. 2050 à 2060, ce sera le moment où nous couperons les arbres- les pins en particulier -que nous allons replanter sur les dizaines de milliers d'hectares aujourd'hui détruits par les flammes.

Il nous faut intégrer des changements inéluctables et profonds aux modèles d'exploitation : choix des essences, diversité des plantations, débroussaillage ou encore lutte contre les parasites. Tout est à remettre à plat et les modèles économiques sont à revoir. Cela ne se limite donc pas

Ma seconde question est donc très simple, monsieur le ministre : allez-vous mettre fin à la suppression constante de postes à l'Office national des forêts, dont la présence déclinante sur le terrain se fait aujourd'hui sentir dans la prévention des incendies et dans la protection de l'environnement ?

et nous avons collectivement la responsabilité de diffuser les consignes et de rappeler la nécessité de lutter contre cette propagation. Reste que les

le dialogue avec l'ensemble des propriétaires de forêts privées, qu'il s'agisse des couloirs de défense incendie ou des réflexions sur les essences. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Notre autonomie énergétique est sérieusement remise en cause. La question du développement de solutions alternatives « urge », tout comme celle de la préservation de nos sols. Voilà un dilemme cornélien que l'agrivoltaïsme peut résoudre, les planètes : production d'électricité par panneaux photovoltaïques inclinables, sur des surfaces tant cultivées que d'élevage, amélioration du revenu des agriculteurs et des productions agricoles, artificialisation maîtrisée des sols.

organise de façon réaliste le développement nécessaire de l'agrivoltaïsme, son accompagnement et son encadrement. Il est clair que l'agriculture doit rester l'activité principale.

Monsieur le ministre, ces installations de panneaux sont démontables, ne présentent aucun danger pour l'environnement et constituent, à l'heure d'un changement climatique galopant, un réel espoir pour nos agriculteurs en matière, d'une part, de protection des cultures et des élevages, d'autre part, d'amélioration de leurs revenus. Comment comptez-vous lever les obstacles et encourager rapidement le développement de l'agrivoltaïsme, pour le bien de nos agriculteurs et de notre souveraineté alimentaire ? La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur

Mme la Première ministre. Depuis presque dix jours, deux gigantesques feux ravagent la Gironde. Cela a été rappelé : plus de 20 000 hectares de végétation ont été brûlés 2 000 sapeurs-pompiers sont mobilisés, appuyés par huit Canadair et deux avions Dash. Je veux, tout d'abord, rendre hommage à ces soldats du feu ainsi qu'aux maires des communes concernées. La Gironde est le département de France où les départs de feux

régulièrement ... Madame la Première ministre, l'État doit rapidement adapter son dispositif de lutte contre les incendies aux évolutions climatiques. Désormais, l'ensemble de la France est concerné : 31 % du territoire métropolitain est boisé.

plus est, les moyens aériens ont fait défaut au début de l'incendie, en particulier à Landiras : le renforcement de la force aérienne nationale de la sécurité civile est urgent, afin que cette dernière puisse agir dès le départ du feu. Outre leur nombre, la localisation des bombardiers d'eau à proximité est primordiale. Face à la rupture majeure que constitue le changement climatique, la prévention est vitale. L'augmentation des départs de feu nécessite un besoin constant en investissement, à la charge notamment

Sur ces deux feux, près de 2 000 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs, ainsi que 200 forestiers, sont engagés. Les moyens aériens déployés à ce jour sont six Canadair et deux Dash. Comme je l'indiquais précédemment, les moyens en renforts nationaux atteignent 1 222 personnes. Comme vous le savez aussi, le Président de la République et le ministre de l'intérieur sont cet après-midi en Gironde, afin de faire le point sur la situation et d'adapter les moyens nécessaires à la lutte contre les incendies en cours. l'État, les collectivités et l'ensemble des forces vives de la Nation se mobilisent pour protéger nos concitoyens et ces territoires, face à des incendies exceptionnels. Madame la ministre, ma question portait sur les actions à venir de l'État. Vous me répondez sur ce qui se passe en détaillant ce que vous avez fait.

Hélas, en l'espace de deux mois, plusieurs meurtres à l'arme blanche vous donnent tort : au mois de mai dernier, un médecin militaire a été tué à Marseille un retraité a été poignardé à Trappes ; le lendemain, une femme a été assassinée à Montpellier ; le 14 juillet, deux jeunes ont été mortellement blessés à Metz et à Amiens. Tout récemment, nous avons tous été extrêmement choqués par un triple meurtre à l'arme blanche à Angers. Trois jeunes hommes, âgés de 16 à 20 ans, issus de la communauté wallisienne, ont en effet été tués alors qu'ils portaient secours à une jeune femme agressée sexuellement. Malheureusement, ces faits se multiplient, et pas seulement dans nos métropoles. Sans réelle stratégie, dans un déni et une émotion « de routine », dirais-je, votre gouvernement participe à la banalisation de cette triste réalité en refusant de nommer ces actes barbares pour ce qu'ils sont, par exemple, de faits divers ou, selon le président Macron, de simples « incivilités ». Monsieur le garde des sceaux, il n'est question ni de stigmatiser ni de prétendre détenir une quelconque baguette magique. Il s'agit simplement de vous interroger sur la réponse que vous apportez aux familles qui ne se résignent pas, qui n'acceptent pas que la vie de quiconque puisse ainsi être aussi facilement fauchée dans la rue.

quelques chiffres, tout aussi dérisoires que les mots, pour affirmer que, depuis de nombreuses années, le nombre de meurtres commis dans ce pays est à peu près stable.

Le quantum moyen en 2000 était de 6 mois ferme : il est aujourd'hui de 9,6 mois, ce qui fait de notre pays l'un des plus sévères d'Europe.

beaucoup de courage et beaucoup de conviction pour restaurer l'autorité républicaine à tous les niveaux, de l'école jusqu'à l'institution judiciaire. Nous comptons sur vous pour le faire. La parole est à M. Denis Bouad, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Comme lui, je tiens à rendre hommage à l'engagement remarquable de nos sapeurs-pompiers et de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Dans les prochaines années, le risque d'incendie sera plus étendu dans le temps, mais également dans l'espace. Les prévisionnistes font état d'une augmentation de 80 % des surfaces brûlées d'ici à 2050.

lutte contre le changement climatique exige des politiques ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, chaque hectare de forêt qui brûle nuit à notre capacité de stocker du carbone.

alors que le risque d'incendie est de plus en plus important, le volontariat de nos sapeurs-pompiers, qui sont seulement rémunérés neuf euros de l'heure, ne pourra à lui seul constituer une réponse sur le long terme. Ma question est donc simple, madame la Première ministre. Alors que les territoires sont différemment touchés par les aléas climatiques, que ce soient par les incendies, les inondations ou la canicule,

les moyens de lutte contre les incendies. J'étais moi-même dans le Gard voilà une dizaine de jours, aux côtés des élus, quand un feu extrême s'est déclaré dans les Cévennes.

les moyens humains et matériels sont considérables : les renforts nationaux marquent la solidarité de tout le territoire pour lutter contre ces feux. Dans ce contexte, monsieur le sénateur, vous attirez l'attention du Gouvernement sur la question, légitime, du financement des SDIS.

par le Gouvernement au Parlement d'ici au 1janvier prochain. Il portera sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. ce rapport devra dresser l'évolution des recettes et dépenses de ces établissements publics, avec des prévisions du court au long terme. Deuxièmement, il fera l'analyse des critères de calcul des dotations et des contributions versées à ces établissements publics et évaluera leur pertinence. Troisièmement, il déterminera les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, pour l'ensemble des financeurs. Il détaillera les conséquences budgétaires propres aux SDIS. Quatrièmement, enfin, le rapport

EDF doit s'engager dans des investissements colossaux : 65 milliards d'euros pour le grand carénage, 90 milliards d'euros pour les EPR (). Le deuxième enjeu est juridique : c'est l'articulation avec le droit européen. Les concessions hydroélectriques sont sous le coup d'un différend vieux de vingt ans avec la Commission européenne ; une quarantaine d'entre elles sont arrivées à échéance. Et que dire du principe du coût marginal, qui lie le prix de l'électricité à celui du gaz ? Il s'agit d'un désavantage pour notre mix

mais il a arrêté la centrale de Fessenheim en 2020 et le projet Astrid en 2019. Sur les concessions hydroélectriques, on a évoqué tout et son contraire : on parlait d'ouverture, de regroupement, de quasi régie. Que d'indécision ! Que de revirements ! Que de retards Aussi, ma question est simple. Au-delà de la nationalisation, monsieur le ministre, comment comptez-vous résoudre les difficultés d'EDF, qui mettent en péril notre souveraineté ?

D'abord, je tiens à dire que je suis toujours très sensible à l'accueil chaleureux que me réservent les sénatrices et les sénateurs. Je remercie le sénateur Gremillet de sa question, qui porte sur des enjeux stratégiques pour notre nation. Le Président de la République a décidé

actuel le plus important pour notre économie et pour notre nation. C'est tardif ! Quelle est la feuille de route qui va être donnée au groupe pour les années qui viennent ? La première urgence est de produire plus, retrouver une capacité de production d'électricité qui soit à la hauteur du groupe. Chacun le voit bien : nous sommes

La deuxième urgence est de réaliser le programme de six nouveaux réacteurs nucléaires qui a été annoncé par le Président de la République au Creusot.

La troisième urgence, énergétique, vous avez parfaitement raison de le souligner, monsieur le sénateur, est de mettre fin à l'absurdité du modèle européen dans lequel le prix de l'énergie décarbonée est aligné sur le prix des énergies fossiles. Nous voulons des résultats rapides sur ce sujet. La présidente de la Commission européenne a commencé à bouger, la commissaire Margrethe Vestager également. Nous voulons réformer le marché européen de l'énergie. Quant à notre stratégie énergétique, elle est très simple. En trois mots, ainsi qu'elle a été rappelée par le Président de République au Creusot : plus de sobriété, plus d'énergies renouvelables et une confiance totale dans l'énergie nucléaire.

Mes chers collègues, EDF, c'est soixante-quinze années d'histoire. N'oublions pas que l'on a légiféré en 1946 pour sa nationalisation ; n'oublions pas que l'on a légiféré en 2004 et en 2010 pour sa modernisation.

Cette mesure est malheureusement déconnectée de toute réflexion sur le devenir d'un secteur en plein bouleversement, Mme Bachelot ayant choisi d'enterrer le débat nécessaire sur la réforme audiovisuelle engagé par son prédécesseur. Elle est également déconnectée du contexte lourd et incertain de nos finances publiques.

Cette mesure redonnerait du pouvoir d'achat aux Français : tel est l'argument. Pourtant, il est question de substituer à la redevance une part de la TVA, laquelle est payée par tout le monde, sans distinction de ressources. Rappelons qu'aujourd'hui 5 millions de foyers sont exonérés de la redevance. Compte tenu des enjeux multiples et complexes, ne serait-il pas sage, comme le réclame l'ensemble d'un secteur très inquiet, de reporter cette décision qui, selon le rapport, n'est pas sans risques juridiques et politiques

la compensation à l'euro près, le versement de l'intégralité des ressources en début d'année pour éviter une régulation en cours d'exercice, une visibilité pluriannuelle accrue du financement.

C'est ce qu'affirment les présidents des entreprises auditionnées la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, selon le scénario choisi, nous savons qu'il y aura un impact sur le budget de l'État et sur la dette publique, dont on nous dit que la « cote d'alerte » est atteinte.

permettant de fédérer l'ensemble des entités affectées par la réforme, offrant une sortie par le haut, ni plus ni moins, aux parlementaires responsables et constructifs. Nous souhaitons ce rapport et ce travail de fond. La parole

Madame la Première ministre, après mon rapport d'information de 2019, qui alertait déjà sur le déclin de la production agricole française, lequel favorise l'entrée toujours plus importante de produits agricoles importés ne respectant pas nos normes après l'épisode du covid, qui nous a fait prendre conscience de notre dépendance à l'égard de produits fabriqués à l'autre bout du monde et qui nous a fait redécouvrir l'intérêt majeur d'une alimentation produite en France

après nous avoir fait croire que vous aviez récemment compris tout cela en nous vantant, par exemple, les bienfaits des clauses miroir et en rebaptisant « ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

sur le modèle qui nous conduit désormais à intégrer des clauses environnementales et sociales dans les accords de nouvelle génération. Je ne doute pas que vous y soyez sensible, monsieur le sénateur. Il prévoit notamment des sanctions commerciales en cas de violation des principaux engagements en la matière. Enfin, c'est un bon accord en ce qu'il protège nos filières agricoles sensibles et soutient nos exportations agricoles et agroalimentaires,

Arrêtons, tant qu'il est encore temps, avec ces injonctions contradictoires ! Nous ne pouvons empiler sans cesse critiques, contraintes et normes, qui tuent la compétitivité de notre agriculture, et la livrer, dans le même temps, à une concurrence déloyale. Vous ne pouvez interdire toujours plus de molécules en France et fermer les yeux sur les produits issus d'une agriculture néo-zélandaise, qui utilise encore de l'atrazine, interdite chez nous depuis 2003 ! Madame la Première ministre,

La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après avoir passé cinq ans à ne prendre aucune décision à la hauteur des enjeux, le Gouvernement est resté muet sur le rôle qu'il entend faire jouer à cette entreprise dans le contexte extrêmement difficile que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur le ministre, quel est votre projet industriel, social et environnemental pour EDF ? Avez-vous renoncé au découpage de l'entreprise, Comment financerez-vous les investissements nécessaires au grand carénage, aux énergies renouvelables et au nucléaire- existant et programmé -, ainsi qu'aux réseaux ? Comment préserverez-vous le caractère public du parc de production hydraulique ? Une OPA va exclure, de fait, les citoyens et le Parlement de ce débat national. Pour donner suite aux intentions, que l'on croyait nouvelles, de dialogue que le Gouvernement affichait voilà quelques jours à peine, allez-vous passer par une loi spécifique ? Nous vous le demandons

À tous ceux qui nous ont expliqué pendant des années que l'on pouvait gagner le combat climatique sans le nucléaire, la réponse est définitive : nous ne pouvons pas gagner la bataille du climat sans reconstruire des capacités nucléaires. Rouvrez Fessenheim ! Je rappelle que le Président de la République est le premier à avoir engagé la réalisation de six nouveaux réacteurs nucléaires et que notre majorité est la première à avoir mis sur pied une université des métiers du nucléaire pour redonner ses lettres de noblesse à l'activité de production d'électricité nucléaire et la première encore à avoir dégagé, au travers de France 2030, des moyens de financement aussi importants pour réfléchir aux réacteurs de petite et de moyenne taille

Nous ne reviendrons pas dessus. Nous voulons marquer, avec la Première ministre, un nouveau départ pour EDF. Cette nationalisation en constitue la première étape. À la direction maintenant, avec l'État, de définir ses priorités. Monsieur le ministre, vous ne répondez pas tout à fait à mes questions. De tergiversations en atermoiements, la France vient de perdre cinq ans. Plutôt dix ! Pour répondre à ses missions de production, EDF doit rester un groupe intégré intégré sous statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Pour l'intérêt national général, nous souhaitons qu'EDF ne soit pas entravée dans son développement. Nous sommes donc favorables à la suppression de l'Arenh, ce qui doit aller de pair

Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. C'est par un décret pris en catimini, au coeur de l'été 2018- le 3 août, précisément -, que le poison a commencé lentement à se répandre. Ce poison, c'est celui de la République des copains,

Depuis lors, madame la ministre, ce poison n'a eu de cesse de miner notre diplomatie, qui pâtit d'une absence de vision, de consultation et de concertation. Depuis le début de l'année, je me suis rendu dans près de trente pays, soit autant de rencontres avec nos postes diplomatiques. Partout, la même inquiétude monte face à une réforme à la fois injuste et incompréhensible. Vous avez pris la décision de supprimer le corps diplomatique. Après cinq ans d'une politique d'improvisation constante, vous avez décidé qu'il était désormais possible de s'improviser aussi diplomate. Or on ne s'improvise pas diplomate : c'est une vocation, une carrière que l'on construit au fil des expériences. Oui, l'inquiétude monte face au manque de considération pour nos diplomates, dont plusieurs dizaines attendent encore leur affectation pour la rentrée. Lorsque vous agissez ainsi, c'est l'image de la France qui est abîmée et la voix de la France qui est affaiblie. Oui, la France peut se targuer de bénéficier d'un solide réseau, qui a su s'ouvrir largement et se diversifier depuis plusieurs années. Oui, la France est riche de ce corps diplomatique, de son savoir-faire et de son expertise respectée partout dans le monde. Et si ce corps doit évoluer, cela doit se faire dans l'écoute, le respect et la concertation, sans esprit partisan, mais certainement pas à travers un décret pris discrètement entre les deux tours de l'élection présidentielle. Madame la ministre, avez-vous conscience de l'image désastreuse que cette réforme injuste renvoie en France comme à l'étranger ? Que comptez-vous faire pour permettre à notre diplomatie de poursuivre sa mission de manière professionnelle et sereine ?

d'Orsay. Je l'expliquerai mieux, en montrant les opportunités qu'elle représente en termes de mobilité interministérielle, en consolidant les garanties obtenues par mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, et en démontrant que quelques contre-vérités n'ont plus lieu de courir. La mise en extinction des corps des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères ne signifie pas, monsieur le sénateur, l'extinction ni des métiers ni des carrières diplomatiques. Le Quai d'Orsay continuera de recruter les meilleurs profils et les diplomates pourront y dérouler des carrières sur la durée. Les amis, oui ! Je compte ensuite examiner la question des missions et des moyens, à la fois budgétaires et en emplois, dans un contexte international où les missions n'ont cessé de croître- climat, santé, biens publics mondiaux, protection des Français ... Enfin, je lancerai une concertation sur l'avenir de notre diplomatie pour réfléchir, notamment avec vous, à l'outil diplomatique dont l'État et les Français ont besoin. Il s'agira d'un exercice important. Nous aurons besoin de vous, de votre regard, de vos idées et de votre exigence pour réussir cette concertation que je souhaite inclusive et positive. La parole

Les 333 salariés licenciés et leurs familles, les habitants et leurs élus se battent depuis des mois contre le démantèlement de l'outil de production et la fuite des savoir-faire de la métallurgie aveyronnaise. Le bassin de Decazeville, par la volonté des collectivités locales, porte en effet un projet industriel réel pour l'avenir de son territoire. MH Industries proposait la reprise du site, avec de véritables perspectives de diversification afin de ne plus dépendre du client unique Renault. Pourquoi l'État n'est-il pas au rendez-vous ? Hier, monsieur le ministre, vous avez déclaré que le repreneur s'était retiré à cause d'une commande insuffisante du client historique et d'une relation client-fournisseur dégradée. dégradée. En tant que représentant de l'État, actionnaire de Renault, vos propos ne sont pas acceptables : l'État serait-il complice d'une quelconque sanction ? Évidemment, vous me répondrez que l'équation économique est peu viable, que l'État et votre prédécesseur ont assuré un suivi constant et que les anciens salariés sont accompagnés dans leur retour à l'emploi ou dans leur reclassement. Monsieur le ministre, ne nous dites pas que les perspectives de réindustrialisation sont bonnes, en particulier en Aveyron : tout un bassin d'emploi souffre et la Mecanic Vallée est fragilisée. Monsieur le ministre, que dites-vous aux élus locaux qui sont désemparés ? Quelles sont vos solutions pour assurer la transition et l'innovation industrielle des fonderies dans les territoires ruraux ?

vous l'avez souligné, la relation dégradée avec le client historique a participé à sa décision, mais aussi et surtout la conjoncture internationale dégradée et le renchérissement des matières premières, qui rendaient l'opération trop risquée à la fois pour SAM et

je suis prêt à travailler avec vous. Très

est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, qui s'est réunie hier, sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observations, je considère ces conclusions comme adoptées.- En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi ordinaire n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable, par dix voix pour et onze voix contre, à la nomination de M. Bruno Lasserre à la présidence de la Commission d'accès aux documents administratifs. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale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

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

Je suis un homme de dialogue et de compromis. Je crois que nous pourrons collectivement parvenir à bâtir des solutions au service de l'intérêt supérieur de la Nation. me semble que cet état d'esprit est aussi celui du Sénat. Je me réjouis donc de pouvoir travailler avec vous sur ce sujet ô combien essentiel pour les Français, la santé. Permettre à chaque Français, quel que soit son revenu ou son lieu de résidence, d'être soigné dans de bonnes conditions redonner du sens au métier de soignant ; sauver l'hôpital ; développer une véritable culture de la prévention : autant de défis majeurs pour lesquels nous aurons besoin de tous, soignants, soignés, élus, pour parvenir à des solutions pragmatiques, efficaces et facilement applicables.

Je le dis avec force, car j'entends et je lis des discours mensongers qui permettent à des commerçants de la désinformation de prospérer sur les réseaux sociaux, et ce au détriment de la santé des Français et de la sauvegarde des valeurs démocratiques.

Le projet de loi qui vous est proposé comprend deux mesures minimales, mais essentielles, pour protéger les Français. En effet, si l'état d'urgence sanitaire est derrière nous, l'épidémie continue. Nous vivons actuellement une septième vague, qui semble être- je reste prudent -sur une phase descendante. Nous connaîtrons sans doute à l'avenir d'autres vagues.

Les dispositions concernées, qui sont simples et proportionnées, ont quatre objectifs : nous permettre de suivre l'évolution de l'épidémie et le nombre de contaminés au jour le jour garantir la libre circulation des personnes, avec l'émission des certificats nécessaires pour se rendre vers des pays qui maintiennent des restrictions ; informer les cas contacts pour qu'ils puissent s'isoler et se tester ; protéger les Français si un variant inquiétant émerge à nos portes. Avant de vous détailler les différentes mesures, je voudrais vous rappeler, comme je l'ai fait lors de mon audition en commission des lois, mon engagement envers les Français et leurs représentants en matière de gestion épidémique. Il est de cinq ordres transparence quant à la situation sanitaire que nous connaissons ; protection de la population par l'adoption de mesures nécessaires pour limiter, autant que faire se peut, la diffusion du virus proportionnalité des mesures adoptées pour que nos concitoyens puissent mener une vie aussi normale que possible ; préservation du système de santé pour éviter le risque de saturation, dans le contexte que nous connaissons et qui justifie pleinement mon engagement aux côtés des professionnels pour l'accès des Français à la santé maintien de la prise en charge des soins hors covid, ce qui est une exigence d'équité vis-à-vis de nos concitoyens. Tout d'abord, conformément à mon engagement de transparence, je voudrais vous communiquer les derniers chiffres dont je dispose sur la septième vague, qui est due aux sous-variants d'Omicron BA4 et BA5. Au 19 juillet, le taux d'incidence s'établit à 1 133 pour 100 000 habitants, en diminution de 16 % sur les sept derniers jours. Il était de 1 433 le 10 juillet. Nous enregistrons en moyenne, sur les sept derniers jours, 95 000 nouveaux cas journaliers.

et 898 personnes sont en soins critiques. Je le rappelle, même si nous semblons être sur la pente descendante de la septième vague, les hospitalisations sont, elles, légèrement décalées dans le temps par rapport à l'évolution des contaminations. La vigilance reste donc de mise. La capacité de l'hôpital à faire face à l'épidémie sera par ailleurs renforcée par l'instruction que j'ai signée voilà une dizaine de jours. Elle traduit la mise en oeuvre des mesures d'urgence de la mission réalisée à la demande de ma prédécesseure Brigitte Bourguignon et entérinée par la Première ministre. Toujours dans mon objectif de transparence à votre égard et pour les Français qui nous écoutent, je veux aussi rappeler notre stratégie face à la covid-19. Elle est claire et peut se résumer en cinq mots prévenir, vacciner, tester, isoler, traiter. Nous devons prévenir la propagation du virus par les gestes barrières. J'appelle ici à la mobilisation citoyenne, car nous ne pourrons pas légiférer à chaque vague de l'épidémie. Les gestes barrières, comme le port du masque en situation de promiscuité, doivent redevenir des réflexes. La vaccination est essentielle. C'est notre arme de protection massive. Je m'insurgerai toujours, en tant que médecin, contre la désinformation qui circule, notamment sur les réseaux sociaux. Le vaccin réduit significativement le risque de développer une forme grave de la covid-19. C'est pourquoi, conformément aux recommandations des autorités scientifiques, nous avons ouvert le deuxième rappel vaccinal aux personnes vulnérables, à savoir les plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées et à risque de forme grave. En cas de doute, test. En cas de test positif, isolement. Dès que nous sommes cas contact ou symptomatiques, nous ne devons pas hésiter. Nous devons réduire les contacts, nous tester, et, si le test est positif, nous isoler jusqu'au rétablissement.

Il existe des traitements curatifs, comme le Paxlovid, qui permettent de diminuer le risque de développer une forme grave de la maladie. Les Français doivent connaître l'existence de tels traitements et pouvoir en discuter avec leurs médecins et pharmaciens. Face à une épidémie qui revient par vague et au risque de l'émergence d'un variant inquiétant, le projet de loi comporte deux dispositions essentielles et minimales.

SI-DEP permet l'enregistrement des tests covid, afin que nous puissions suivre l'épidémie. C'est également grâce à ce système que nous produisons les certificats permettant à nos concitoyens de voyager vers des pays qui ont maintenu des restrictions sanitaires à l'entrée Je me félicite que la commission des lois du Sénat ait prolongé, en cohérence avec le règlement européen, la validité de SI-DEP jusqu'au 30 juin 2023. Cela garantira aux Français la possibilité de voyager en Europe et dans le monde, en leur permettant de disposer des certificats de test ou de rétablissement que tout État peut exiger pour entrer sur son territoire. Il s'agit d'une évolution bienvenue. Nous conserverons ce thermomètre irremplaçable de l'épidémie jusqu'à cette date. Contact Covid nous permet d'identifier les cas contacts, de les informer et de les protéger. La commission des lois a maintenu, pour ce qui concerne ce système d'information, la date du 31 janvier, qui avait également fait consensus à l'Assemblée nationale. L'article 2 a connu un destin mouvementé. Dans sa version initiale, il nous offrait la possibilité, comme c'est le cas dans le droit en vigueur depuis plus d'un an, de demander certains justificatifs aux personnes qui se déplacent depuis ou vers le territoire hexagonal. Je pense en particulier à la Corse et aux collectivités d'outre-mer.

Je me félicite que la commission des lois ait confirmé le principe de l'intérêt d'une telle disposition. Je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu. tel travail peut, je le crois, être poursuivi dans cet hémicycle sur quelques points d'importance, pour donner sa pleine mesure à l'article. Je soutiendrai certains des amendements qui ont été déposés pour contribuer à améliorer encore, avec vous, le texte adopté par la commission des lois. la commission des lois. Cette dernière a également souhaité supprimer formellement, au lieu de simplement laisser les dispositions s'éteindre, le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire. Si cela allait sans dire, cela va peut-être mieux en le disant. Le Gouvernement, qui avait suivi l'avis du Conseil d'État sur ce point, comprend la préférence de votre commission pour une suppression plus nette, même si cela suppose des travaux légistiques un peu sophistiqués. Enfin, vous avez souhaité préciser le contenu du rapport prévu à l'article 3, afin qu'il aborde les potentielles dispositions de droit commun qui seraient pertinentes face aux menaces sanitaires, en lieu et place d'un régime d'exception. Le Gouvernement répondra à cette demande d'information.

de respecter les gestes barrières et de porter le masque dans le métro. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'obligation qu'il faut faire preuve de négligence

nous réjouir d'entrer dans une période où le retour de la liberté sera acté par le Parlement, sans retour possible aux pouvoirs d'exception que nous avions consentis tout en les proportionnant strictement aux exigences de la situation sanitaire. L'épidémie n'est pas terminée. Hier encore, il y a eu 130 000 cas de contamination avérés, et certainement beaucoup d'autres qui n'ont pas fait l'objet de test.

la courbe d'évolution de l'épidémie évoque de manière assez nette, selon les épidémiologistes, celle de toutes les épidémies virales

Allemagne et un million aux États-Unis. Si on rapporte le nombre de décès à la population, nous ne sommes pas un pays spécialement performant

démontrant l'inutilité de ces derniers, à l'absence de gel hydroalcoolique et à la nécessité, faute de moyens de lutter efficacement contre l'épidémie, d'un confinement qui, lui, a été extrêmement efficace pour donner un coup d'arrêt aux contaminations par le premier variant du virus. En songeant à toutes les victimes

que nous aurions été spécialement mauvais dans la lutte contre le covid. La réalité se situe quelque part entre les deux. Au Sénat, nous aurions aimé que la France

simplement voulu établir un texte simple et clair, en sortant d'un entre-deux qui nourrissait le soupçon.

pour la réintégration des personnels suspendus- je dis bien « suspendus », et non pas « licenciés » -parce qu'ils ne voulaient pas respecter l'obligation vaccinale qui leur était imposée dans l'intérêt des malades ou des personnes prises en charge dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Ces trois choses toutes simples sont bien dans l'esprit du Sénat. Elles sont en cohérence avec ce que nous avons toujours fait. En responsabilité, nous sommes prêts à accepter de prendre des mesures de protection, mais celles-ci doivent être strictement proportionnées aux exigences de la situation et ne peuvent être mises en oeuvre que sous le contrôle du Parlement. J'évoquerai tout

qu'il faut être clair ! Nous voulons abroger l'état d'urgence sanitaire pour que l'on ne puisse plus y revenir. Nous voulons abroger le régime de gestion de la crise sanitaire, qui s'est ajouté à l'état d'urgence sanitaire. Vous pensez que les choses vont sans le dire. Nous vous répondons, selon l'usage, qu'elles vont encore mieux en le disant et, en l'occurrence, en l'écrivant pour le graver dans le marbre de la loi. En effet, il est trop facile d'ouvrir le code de la santé publique au mois d'août et de constater que l'état d'urgence y figure encore. Si, un jour, nous avons une nouvelle épidémie, nous voulons que vous reveniez ici et que vous discutiez pied à pied tous les pouvoirs que vous réclamerez au Parlement. Nous ne voulons pas que vous vous contentiez d'une ligne visant à rétablir l'état d'urgence sanitaire.

que le Gouvernement peut prendre un décret à sa discrétion : il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais ces personnels n'ont pas été licenciés ; ils ont seulement été suspendus. La suspension ne peut pas durer au-delà des nécessités médicales ; elle est faite pour protéger les malades, les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous exigeons

Ces dernières années nous ont montré que quelques sophismes pouvaient avoir bien trop facilement la peau de nos principes et de nos libertés fondamentales. Je vous invite à relire Saint-Augustin d'Hippone : « À force de À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Au mois de juillet 2021, je m'opposais ici avec vigueur à l'instauration du premier passe sanitaire de l'histoire de notre pays. Vous aviez alors été nombreux, nombreux, mes chers collègues, à vouloir couler les arguments de la raison sous l'argument d'autorité selon lequel la charge virale du variant delta était « mille fois plus élevée que celle du précédent variant C'est surtout le ridicule de certains qui a été multiplié par mille ! Ce passe sanitaire, qui est avant tout un passe vaccinal, était déjà disproportionné. Un an après, j'y reste totalement opposé, car il faut un peu de constance. Après avoir voté ce passe vaccinal, notre collègue Bruno Retailleau n'a pas rougi lorsqu'il a déclaré récemment : « Le passe n'a aidé en rien dans la lutte contre le covid. » C'est ce que nous disions à l'époque, dès l'instauration du passe. Au mieux, on nous a ri au nez ; au pire, on nous a accusés de mettre la santé des Français S'il n'est jamais trop tard pour confesser ses erreurs, votre inconstance a des conséquences graves, car elle instaure des précédents. Il faut en finir avec cette honteuse culpabilisation infligée aux Français, qui les désignait responsables de la saturation hospitalière. L'hôpital s'effondre parce que vous avez sacrifié durant des décennies la rigueur sanitaire au profit de la rigueur budgétaire ! Il s'effondre parce que vous avez suspendu les soignants ! Il s'effondre parce que vous avez fermé des milliers de lits, y compris en période de covid ! Il s'effondre parce que vous y accueillez le monde entier Le texte du Sénat perpétue une rupture d'égalité entre les citoyens français, en maintenant le passe sanitaire entre la métropole et les territoires ultramarins. De plus, vous imposez un passe sanitaire aux enfants mineurs à partir de 12 ans, alors que cette mention n'existait plus. C'est totalement injustifié. Votre texte perpétue les systèmes d'information liés au covid jusqu'en mars 2023. De prolongation en prolongation, cette mesure d'urgence est en voie de pérennisation, malgré les dangers liés à la protection des données sensibles, qui sont collectées, alors que de nombreuses failles de sécurité ont pourtant été relevées. Alors que la France est un coupe-gorge, alors que la France brûle, alors que l'hôpital s'effondre, ce texte du Sénat ne répond toujours pas à l'impératif de la réintégration de 15 000 soignants, pompiers et forces de l'ordre ! Vous qui les avez suspendus sans délai, vous refusez de les réintégrer immédiatement en vous déchargeant, bien sûr, de

et la possibilité pour l'exécutif, en cas de nécessité, d'instaurer un passe sanitaire lors de déplacements hors de l'Hexagone ou à l'international. S'il s'agit d'une étape supplémentaire vers la fin de l'état d'urgence sanitaire, des mesures exceptionnelles pourront toujours être prises par l'exécutif, contrairement à ce que proclament- nous y reviendrons lors de l'examen des amendements

Mais nous nous sommes toujours opposés aux mesures que nous jugions inutilement coercitives, au perpétuel état d'exception au sein duquel nous devions légiférer, aux volontés de l'exécutif d'escamoter le débat parlementaire, voire d'ignorer la représentation nationale. Jusqu'à présent, nous partagions ces principes avec la majorité sénatoriale. Mais M. le rapporteur semble faire volte-face, notamment sur le vaccin. Pas du tout ! Peut-être est-il plus préoccupé par la conciliation des différentes sensibilités de sa formation politique que par la cohérence des positions du Sénat Nous n'avons pas fait grand-chose en commission des lois », a-t-il affirmé avec son goût de la litote. Ce n'est évidemment pas exact. La commission a décidé, à rebours des positions constantes du Sénat, de retirer le justificatif de statut vaccinal du passe sanitaire aux frontières

collègue Bruno Retailleau a déclaré le 7 juillet 2021 : « Nous sommes favorables à cette vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger ceux qui viennent se faire soigner. » se faire soigner. » « Cette obligation vaccinale contre la covid-19 participe du devoir d'exemplarité, mais aussi du devoir éthique qu'ont les soignants de ne pas nuire et de protéger les personnes vulnérables

parfois ! Vous avez également proposé la prorogation du système SI-DEP. Pour notre part, nous considérons que tout doit être calé au 31 janvier 2023.

nous connaissons une évolution favorable de la pandémie, qui, aujourd'hui, présente un caractère peu générateur de suites mortelles ou graves.

Ce bilan devra être réalisé de manière pluraliste et approfondie. Car il faut, certes, tourner la page des mesures contraignantes, mais il faut aussi apprécier

de faire figurer dans le code de la santé publique, dont c'est quand même une des finalités premières, l'éventail des mesures contraignantes. Par nature, ces mesures supposent une base législative

mais sur la base d'un travail approfondi. J'ajoute que ce débat de bilan d'efficacité pluraliste pourrait être utilement complété par une demande d'avis du Gouvernement au Conseil d'État, lequel est spécialement accoutumé à se prononcer sur le bon équilibre entre des mesures de contrainte et un dispositif de protection des libertés en cas de situations d'exception. Je fais remarquer, d'ailleurs, avec un tout petit peu de malice, que nous légiférons dans le délai du 31 juillet et que, ici même, le choix de ce délai avait été assez discuté. La période que nous venons de vivre et l'observation que nous faisons du débat à l'Assemblée nationale, dans un contexte postélectoral encore assez animé, montre qu'il n'aurait sans doute pas été très sage d'avoir à légiférer en pleine campagne présidentielle. Le Gouvernement a introduit dans son projet deux mesures principales qui sont des mesures à l'effet très limité et très modéré de prévention de la pandémie : le maintien du système d'information, qui qui doit identifier les mouvements de contamination et avertir les personnes intéressées ; une identification et une prévention des risques liés aux mouvements transfrontières ou transcontinentaux, y compris sur le territoire français avec les outre-mer et la Corse.

savoir celle des personnels de santé, mais aussi des autres personnels de contact, suspendus du fait de leur refus d'appliquer une obligation vaccinale, laquelle correspondait à un intérêt public et sanitaire évident.

la décision de levée de l'obligation vaccinale peut être prise de façon différenciée suivant les catégories professionnelles. Entre les soignants directement au contact des malades et d'autres personnels-

Cela a baissé nettement- vous l'avez indiqué, monsieur le ministre -, même si le nombre d'hospitalisations augmente, car il y a un décalage. La saison d'été est favorable, mais l'avenir est toujours très incertain. Nous avons examiné plusieurs textes

à ne pas être à rebours de son évolution. De plus, nous apprenons l'existence d'un variant Centaure, plus contagieux et plus grave, qui, comme dans la mythologie, développe de nombreux successeurs Le projet de loi permet de maintenir deux mesures essentielles pour un contrôle de l'évolution des contaminations. La première, qui a été conservée, consiste à proroger les systèmes informatiques qui assurent un suivi des contaminations a été rejetée par l'Assemblée nationale, consistait à maintenir la présentation du passe sanitaire pour limiter la propagation du virus lors des déplacements.

et Territoires considère que le contrôle de la propagation du virus est utile pour nos concitoyens, pour les hôpitaux où le personnel a été tellement sollicité, ainsi que pour l'ensemble de notre pays. Il soutient donc le rétablissement de l'article 2. Mais il souhaite que figure également la possibilité pour les voyageurs de présenter soit un test négatif, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat de vaccination. Certes, la vaccination n'apporte pas une garantie complète contre la contamination,

La commission des lois a par ailleurs ajouté la possibilité de réintégrer les soignants qui ne seraient pas vaccinés dans l'hôpital, dans les Ehpad, dans les établissements médicaux sociaux, ainsi que dans les services Monsieur le rapporteur Philippe Bas, je ne nie pas votre expertise. Elle n'est pas médicale ! Vous avez notamment été un excellent ministre de la santé de Jacques Chirac.

que l'État, éclairé par les scientifiques, décide de la réintégration des personnels soignants non vaccinés dans le cadre de la protection des patients et du personnel de soin.

Permettez-moi cependant d'observer que, d'un texte technique de deux articles, portant pour moitié sur les conditions d'accès au territoire national, nous sommes bien revenus à des sujets très sanitaires. Parmi nos concitoyens, la fatigue des vagues successives de la pandémie de covid-19 est de plus en plus perceptible et fait désormais place à une sorte d'indifférence, quand il ne s'agit pas d'un rejet pur et simple des mesures de gestion le sais, sur ces travées, l'accumulation de textes ne réjouit pas davantage. Pour autant, nous ne pouvons que constater que l'épidémie perdure et s'est installée dans notre quotidien. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre de désarmer. Si nous avons tous envie d'en finir avec le virus, nous ne l'abolirons pas par voie législative. Le Gouvernement lui-même a cependant donné le ton avec un texte minimaliste qui comprend, d'une part, le SI-DEP, thermomètre de l'épidémie dont il serait tout de même difficile de se passer,

Face à l'épidémie et aux orientations données par le Gouvernement, le Sénat a toujours eu une attitude responsable, monsieur le ministre. Aujourd'hui, le Gouvernement fixe un cap différent. La responsabilité nous oblige à regarder aussi ce que le texte ne contient pas. Je ne parle pas ici d'un énième comité, laissant croire que la direction générale de la santé, le Haut Conseil de la santé publique ou encore Santé publique France auraient disparu dans notre pays. Je veux plutôt parler de la protection des plus fragiles, ainsi que de la protection de l'hôpital et des établissements médico-sociaux en particulier. C'est pour eux que nous avons consenti tous ces efforts ; ne l'oublions pas Au 1 août, il n'y aura plus de passe sanitaire à l'hôpital ou dans les Ehpad, et la disposition légale permettant aux chefs d'établissement d'imposer le port du masque à l'hôpital, dans les Ehpad, dans les cabinets médicaux, sera caduque. Comment justifiez-vous la levée de ces mesures, monsieur le ministre ? C'est cette même idée qui avait conduit la commission des affaires sociales à soutenir voilà un an l'obligation vaccinale de personnes travaillant auprès de personnes vulnérables, au nom de l'éthique des soignants et de l'exemplarité. La suspension de l'obligation vaccinale n'est pas la solution magique à la pénurie de personnel à l'hôpital, qui a bien d'autres causes ; nous le savons tous ! Mais le Président de la République a évoqué une telle possibilité au mois de juin. Et vous-même, monsieur le ministre, avez considéré devant la commission des lois

un dernier mot sur la méthode. Au début de la crise, la base donnée par le code de la santé publique a été considérée comme trop fragile et il a fallu construire un dispositif juridique spécifique. Dont acte. C'est ce qui nous a valu une avalanche de textes ; nous examinons le dernier aujourd'hui. Au fil de ces textes, le Gouvernement nous a habitués à insérer des amendements sur des mesures de gestion qu'il pouvait tout à fait anticiper, comme la garantie de financement des hôpitaux. Je constate depuis peu qu'un simple arrêté ministériel prévoit, par exemple, la prise en charge à 100 % des téléconsultations, qui figurait dans deux précédentes lois d'urgence. Que faut-il attendre demain ? Vous prenez désormais des arrêtés ministériels sur ce même fondement juridique, jugé fragile par le Conseil d'État. Si les amendements déposés ne nous conviennent pas, sachez que les dérogations à la loi par simple arrêté nous déplaisent encore plus.

? Pourquoi n'inscrivez-vous pas certaines dispositions aujourd'hui dans le texte ? Que comptez-vous faire concernant le financement des hôpitaux, alors que la garantie a cessé au 30 juin dernier ? Sur le fond du texte, alors que le Gouvernement agit désormais par voie réglementaire, je suivrai les orientations définies par la commission des lois. Pour le reste,

Le Gouvernement vient donc vers nous pour permettre le maintien de dispositifs liés aux données personnelles de santé covid et la possibilité d'établir de nouveau un passe aux frontières. Tout d'abord, je tiens à saluer votre présence, monsieur le ministre de la santé ; cela nous change de votre prédécesseur

Nous avons maintes fois exprimé nos regrets d'avoir, comme l'ensemble du pays, subi les décisions solitaires et tardives du Président de la République. Puisque nous avons commencé une nouvelle ère de discussion et de compromis- mais pas avec tout le monde .... -, je souhaite renouveler auprès de cette nouvelle équipe gouvernementale toutes les raisons de nos inquiétudes et toutes les propositions que nous souhaiterions vous convaincre d'adopter.

L'article 2, réécrit par la majorité sénatoriale, reste trop problématique à nos yeux. Certes, il limite la présentation d'un certificat de voyage aux personnes venant de l'étranger sur le sol français en cas d'apparition d'un nouveau variant présentant une menace grave, ou à toute personne souhaitant se rendre dans les collectivités ultramarines en cas de risque de saturation hospitalière sur place. Mais il maintient cette obligation dès l'âge de 12 ans. Si nous saluons le fait que le rapporteur ait prévu une clause de revoyure devant le parlement, la codécision qui devrait être inhérente à toute modification significative à toute modification significative des libertés, telle que celle d'aller et de venir, doit se faire de manière- je le redis -concertée, mais surtout éclairée et précise. Éclairée, d'abord. Le Parlement doit bénéficier des mêmes informations que l'exécutif. Il est regrettable, pour ne pas dire plus, que nous ne soyons pas destinataires de manière concomitante au Gouvernement ou au Président de la République des travaux du Conseil scientifique. Je pense par exemple

santé est atteinte. Les autres mesures de veille et de sécurité sanitaire brillent par leur absence. Nous avions, bien avant le Gouvernement, engagé la discussion sur la troisième dose. Nous l'avions alerté sur les disparités vaccinales, en lui demandant de s'attacher à comprendre et à combattre de tels déséquilibres. Que dire sur la première mesure face à un virus qui circule dans l'air ? Toujours aucune action du Gouvernement concernant l'encadrement des prix des FFP2 ! Toujours aucun plan ou mesures solides sur l'air dans les lieux fermés, comme les écoles, dont la sécurisation doit être votre priorité

Nous, sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, restons persuadés qu'il est urgent d'aider les Français à s'habituer au fameux « vivre avec », mais pas à n'importe quel coût. Tout cela doit se faire de manière sécurisée et généralisée. Nous attendions des mesures fortes dès maintenant pour aller vers les populations non vaccinées, des mesures claires sur le prix des masques efficaces comme les FFP2, sur la gratuité des tests de dépistage, point essentiel pour ne pas faire des Ultramarins et des Français de l'étranger des citoyens de seconde zone. des rappels forts de l'importance des mesures barrières pour ne pas transformer le vaccin en un outil à l'effet pervers. Nous souhaitions des discussions éclairées sur la nécessité ou l'absence de nécessité de conserver les données en jeu dans l'article 1. Nous attendions des actes et un accompagnement financier sur la qualité de l'air dans nos écoles, maintes fois repoussés et promis par le Président de la République alors en campagne. Enfin, nous espérions un dialogue réel sur les dangers connus, les dangers prévisibles et les retours d'expérience de la gestion de ces deux dernières années. Rien de

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite d'abord réitérer notre soutien à l'ensemble des personnels de santé et paramédicaux, qui prennent en charge depuis deux ans les patients de la covid-19 malgré les erreurs stratégiques du Gouvernement, les mensonges, les insuffisances de masques, de tests, de vaccins, de purificateurs d'air, ... Eh oui ! ... Et qui subissent désormais les démissions des professionnels lassés de travailler dans des conditions indignes pour les patients et pour eux-mêmes. Ce onzième projet de loi sanitaire, en raison du rebond de l'épidémie de covid-19 et du sous-variant BA5, interroge sur la volonté réelle du Gouvernement d'investir dans notre système de santé pour se doter des capacités de prise en charge des malades. la fin du mois de mai, les 120 services d'urgence en détresse sont rejoints désormais par 13 autres. Depuis 2017, 17 000 lits d'hospitalisation ont été fermés, dont 5 700 en pleine pandémie. pandémie. Près de 100 000 postes sont vacants à l'hôpital. Et, malgré tout cela, le Gouvernement refuse la réintégration des personnels suspendus, alors même que les études internationales démontrent que si la vaccination joue un rôle dans la diminution de la transmission du virus, d'autres stratégies sont aussi, voire plus importantes. Je pense à la mise en place de capteurs de dioxyde de carbone, à l'installation de purificateurs d'air dans les lieux clos et au respect des gestes barrières. C'est la raison pour laquelle notre groupe a déposé un amendement visant à réintégrer les personnels de santé et les pompiers suspendus. Avec ce premier texte, le Gouvernement a découvert la réalité du Parlement. À cet égard, la suppression de l'article 2 à l'Assemblée nationale a rappelé au Gouvernement, qui ne dispose pas d'une majorité absolue, la nécessité d'écouter les autres forces politiques, ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'ici. Le Le rapporteur de la commission des lois a modifié le texte en rétablissant les dispositions supprimées à l'Assemblée nationale tout en essayant de les encadrer davantage pour leur donner un caractère plus acceptable. Comment ne pas pressentir- je vais être quelque peu impertinente -une entente entre Les Républicains et le Gouvernement, dont le terrain serait le projet de loi sanitaire et le texte sur le pouvoir d'achat ? Nous serons très attentifs, monsieur le rapporteur, à l'attitude de la majorité sénatoriale. Allez-vous céder, notre genre ! ... en échange de je ne sais quel arrangement ? Ou bien, allez-vous tenir bon ? Il faut reconnaître que le maintien d'un dispositif d'exception du Gouvernement et le respect des libertés de nos concitoyens relevaient d'un exercice d'équilibriste. Notre groupe rappelle sa constance sur le refus des dispositifs d'exception et du passe sanitaire. Nous l'avons toujours dit, l'efficacité de la lutte contre la pandémie passe évidemment par la vaccination. Mais elle réside également dans la force de notre système de santé, dans les moyens donnés au service public- je pense à l'école -et dans le respect des gestes barrières, par une information régulière, permanente, accessible. Il est singulier que la seule réponse soit encore et toujours la coercition, et non une nouvelle politique de santé. Pour notre groupe, il est également plus que temps de mettre fin aux systèmes d'information qui permettent la levée du secret médical et au stockage des données personnelles médicales. L'évocation d'un risque pour nos concitoyens de ne plus pouvoir voyager en Europe si notre Parlement ne votait pas la prolongation de tels systèmes d'exploitation, alors que la liberté de circulation des personnes en Europe a été préservée même au plus fort de la pandémie, ne peut pas s'entendre. Elle se limite à la sphère technocratique, alors que la préservation des données est une question hautement politique, qui doit se régler à l'échelon européen également. M. Macron s'y est-il intéressé lors de sa présidence de l'Europe ? Enfin, la possibilité pour le Gouvernement de rétablir un certificat sanitaire de voyage pour les déplacements à destination ou en provenance de la Corse ou d'une collectivité ultramarine nous apparaît comme un très mauvais signal envoyé à nos concitoyens. La rédaction de la commission est, certes, plus acceptable que celle du Gouvernement, mais nous considérons pour notre part qu'il serait préférable d'instaurer un droit d'initiative de cette mesure pour les élus ultramarins, et non une simple consultation. Le Gouvernement serait bien avisé de lancer un plan d'investissement des services de santé ultramarins pour rattraper le retard accumulé depuis des années. La levée des sanctions contre les soignants est là-bas d'une très grande urgence. L'envoi de forces répressives, plutôt que de moyens pour la santé, y a été très mal vécu. En conclusion, par cohérence avec l'opposition que nous avons exprimée dès les premiers jours à l'instauration du passe sanitaire et du passe vaccinal, et en l'absence de dispositifs visant à renforcer notre service public de santé, en l'absence de gratuité des tests, en l'absence de fourniture de masques FFP2 aux personnels médico-sociaux, en l'absence pour la rentrée scolaire prochaine de purificateurs d'air et de capteurs de CO2 dans les écoles, le groupe CRCE votera contre ce projet de loi. Certes, le travail de la commission des lois du Sénat atténue le texte gouvernemental, mais il n'annonce ni de près ni de loin un changement de politique sanitaire. La parole est

chers collègues, après plus de deux années de productions législatives dédiées à la gestion de la crise sanitaire, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est-il le dernier ? Nous l'espérons sincèrement. Nous avons en effet vécu depuis 2015 sous des régimes d'état d'urgence successifs, les trois premiers du fait de l'urgence liée au risque terroriste, les suivants, puis

trois options s'offrent au Gouvernement : premièrement, ne rien faire et laisser s'éteindre- dans quelques jours, donc -les dispositions de gestion de crise, dont j'ai souligné en préambule le caractère exorbitant ; deuxièmement, demander au Parlement de renouveler

collectivement un travail collaboratif efficace, car notre système de santé aura besoin de toutes les forces. C'est le treizième texte sanitaire que nous examinons depuis le début de l'épidémie de covid-19. Si un régime d'exception a très tôt été mis en place pour lutter plus vite et plus efficacement contre le virus, les parlementaires ont aussi été consultés à de très nombreuses reprises par le Gouvernement pour porter la voix des citoyens des élus locaux, dont la vie et le travail ont été profondément bouleversés depuis plus de deux ans. Ce nouveau projet de loi acte la fin des régimes d'exception, et donc de l'état d'urgence sanitaire au 31 juillet. Contrairement à ce que certains ont laissé croire ces derniers jours, il est question non pas de prolonger l'état d'urgence, mais de prévoir un système de veille et de garde-fou pour continuer à lutter contre cette épidémie, qui est loin d'être achevée, même si la situation est en voie d'amélioration ; il faut aussi le reconnaître,

la covid prend une trajectoire de virus plus classique. Mais les populations les plus à risque doivent toujours être protégées, tout comme nos hôpitaux et l'ensemble de notre système de santé, qui se trouvent structurellement en situation de surchauffe. Il reste donc prudent de maintenir un système de veille, tout en faisant le maximum pour reprendre une vie normale. Afin d'être réactif en cas de survenue d'un variant plus virulent, le projet de loi prévoit un contrôle de l'épidémie aux frontières et les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid. Nous ne présenterons pas d'amendement sur l'article 1, convaincus de la nécessité de prolonger ces deux systèmes, qui permettent de suivre l'évolution de l'épidémie. Par ailleurs, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait à l'avenir envisager d'utiliser plus finement ce type de données pour gérer les consignes sur des territoires plus ciblés, en fonction de l'évolution des contaminations sur le terrain. Les choses sont plus complexes concernant l'article 2, qui offre la possibilité au Gouvernement, en cas de résurgence de l'épidémie, de freiner les déplacements aux frontières. Nous sommes en effet circonspects sur la création d'un « certificat de voyage » nécessitant un simple test de dépistage virologique. Le passe sanitaire existe depuis maintenant plus d'un an. Il est connu et

? Il faut le dire, il n'est pas vrai que le vaccin ne limite pas la circulation virale, même s'il ne la limite effectivement pas complètement. Nombreuses sont les études qui prouvent combien le vaccin a réduit la contagiosité.

et compris à nos concitoyens. Telle est la position qui sera défendue par mon groupe, en préférant le passe sanitaire au certificat de voyage. J'en viens à la suspension des soignants non vaccinés. Nous considérons que l'article 2 introduit une ambiguïté. La loi actuelle prévoit déjà la possibilité, sur avis de la Haute Autorité de santé, de supprimer l'obligation vaccinale contre la covid-19 en cas d'amélioration significative de la situation épidémiologique. Ce nouvel article adopté en commission peut être perçu comme une réintroduction des soignants suspendus.

Au-delà du caractère anecdotique de l'effet de ces suspensions sur le système de soins- on parle de 0,4 % à 0,5 % des effectifs nationaux -, nous devons être fermes et clairs sur les valeurs de civisme et d'exemplarité,

opposition, et un gouvernement butant sur la conciliation. Ce serait un tort de penser que le Sénat deviendrait l'antichambre de l'exécutif. Ces deux dernières années, cet hémicycle a connu de longs débats animés, qui ont parfois eu des retombées importantes sur la vie des Français. Dans le cadre du projet de loi, une tâche difficile nous incombe : trouver le juste milieu, conciliant liberté et sécurité avec l'impératif de santé publique. Pourtant, l'exécutif s'obstine à tout prix à instaurer un régime transitoire à l'état d'urgence sanitaire. À l'origine, celui-ci devait durer jusqu'au 31 mars 2023. En commission, il a été jugé pertinent de s'aligner sur les réglementations européennes et de reporter cette date au 30 juin 2023. En d'autres termes, pour voyager librement partout, la présentation d'un certificat numérique covid sera encore nécessaire. Permettez-moi de m'interroger sur les bienfaits d'une telle prorogation. Alors que nous pensions en finir avec l'état d'urgence sanitaire, nous devons à présent composer avec avec un régime transitoire aux contours encore incertains. Le Gouvernement a encore failli à la mission de transparence qui lui incombe en proposant un texte resserré manquant de clarté. Il n'en demeure pas moins que nous mettons officiellement fin au régime de l'exception. Les risques d'un passe sanitaire, d'un couvre-feu ou d'un potentiel confinement sont définitivement exclus. Au fil de l'épidémie, nous nous sommes adaptés tant bien que mal aux mesures prises par le Gouvernement. Celles-ci, qui ont considérablement divisé les Français. Une réelle fracture s'est créée au sein de la société entre vaccinés et anti-vaccins. Toutefois, la réécriture proposée par le Sénat préconise la présentation d'un certificat sanitaire de voyage pour les territoires ultramarins en cas de saturation des systèmes de santé locaux, et après consultation des exécutifs et parlementaires locaux. Il est essentiel de réfléchir à terme Le réchauffement climatique entraînera inévitablement de nouveaux risques sanitaires du même genre. je vous remercie

Plus de 150 000 Français en sont décédés, dont 25 000 depuis le début de l'année. Avec le temps, les mesures que nous devons adopter évoluent. Dans Dans son projet de loi, le Gouvernement estime nécessaire de maintenir le système de surveillance épidémiologique et de prévoir l'hypothèse de restauration de contrôles pour les déplacements au-delà de l'Hexagone. Ces deux demandes nous paraissent justifiées, et nous les approuverons, sous réserve de quelques précisions. Mais la pandémie n'est pas finie, et nous attendions de ce texte qu'il exprime la vision du Gouvernement sur les grands axes : maintien d'une protection collective large par la vaccination ; dispositif assurant la qualité de l'air des lieux clos clos ; pédagogie sur le port du masque dans les lieux clos, en particulier pendant la saison hivernale. Car nous devons prévoir, anticiper les évolutions possibles pour les prochains mois, ainsi que nous y invite à raison le Conseil scientifique dans son dernier avis. Sortir de l'état d'urgence sanitaire, sortir des mesures d'exception, ce n'est pas sortir de la pandémie. Nous n'avons aucune gloire à tirer de l'abandon de mesures devenues inutiles : cela ne fabrique aucune mesure utile pour la suite d'une pandémie qui se poursuit. Or nous devons nous contenter d'un texte réduit au minimum, qui, après sa réécriture par la commission des lois, esquive toujours des sujets importants, voire les a écartés. Dans quelques jours, le Conseil scientifique sera dissous et aucune indication n'est avancée sur un dispositif efficace de veille, d'alerte et de propositions en cas de nouvelle crise. Le nouveau dispositif ne saurait trop tarder, monsieur le ministre. la pandémie n'est pas finie. La commission des lois a procédé à un salutaire toilettage du code de la santé publique, mais en nous ramenant à l'état crise de la législation ; nous sommes au milieu du gué. Il nous faudra rapidement avancer pour définir un nouveau cadre adapté. Malheureusement, en introduisant dans le projet de loi, au terme de son mémorandum, la question de la réintégration des soignants non vaccinés, la commission prend une position politique que nous ne partageons pas.

Nous sommes ici, sur ce premier texte d'une nouvelle législature, pour montrer que le compromis auquel nous appellent les Français doit se fonder sur un partage commun de ce qui est juste pour notre pays, et non sur des messages envoyés aux plus extrémistes et aux populistes. Le vaccin est une chance pour la santé publique. Il a sauvé, il sauve et il sauvera tant de vies. Nous le défendons- il ne doit pas disparaître de l'article 2 ! -, comme nous défendons l'idée que le métier de soignant ne s'exerce que dans l'acceptation des règles de protection réciproque et collective. Se soustraire à ces règles, c'est renier une part de l'éthique et de la grandeur des professions concernées. Tant que l'on ne les accepte pas, c'est un aller sans retour. Alors, laissez les 0,3 % qui refusent la règle commune là où ils sont, et nous exprimerons ainsi soutien et compréhension envers l'immense majorité des soignants. Car si nous exonérons cette infime minorité de ses obligations, nous récolterons incompréhension et colère dans nos hôpitaux, nos cabinets médicaux et nos Ehpad. Ehpad. Tel est notre état d'esprit, celui d'un travail parlementaire engagé pour mieux anticiper nos réponses à l'épidémie, et pour répondre avant tout au devoir de protection de nos compatriotes. La parole

Consacré cette fois-ci à la « veille et à la sécurité sanitaire », il diffère toutefois fortement des précédents, tant par son contexte que par son contenu. Le contexte, nous le connaissons évidemment tous. Il est d'abord sanitaire. Nous faisons face à une septième vague qui se répand rapidement, mais qui- c'est heureux ! -aura été moins virulente que les premières et qui semble fortement décliner depuis une semaine. Comme le rapporteur, Philippe Bas, a pu le souligner précédemment, l'évolution de la pandémie est cohérente par rapport à ce que nous observons pour d'autres virus, mais elle ne doit pas être ignorée pour autant. Il y a aussi un contexte politique que nous connaissons, et sur lequel je ne m'attarderai pas. Enfin, il y a le contexte juridique. Plus de deux ans après l'adoption de la première loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la France est sur le point de sortir de l'essentiel des régimes dérogatoires du droit commun institués pour la gestion de cette crise sans précédent. C'est l'une des raisons pour lesquelles la commission a suivi son rapporteur et changé le titre du texte. Ce dernier reflète désormais la réalité J'en viens au contenu du projet de loi. C'est un texte court, pas seulement technique, comme initialement annoncé, mais avec des enjeux politiques. Il était initialement proposé au législateur de maintenir seulement deux dispositifs de veille sanitaire : d'une part, les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid, afin de permettre aux autorités de santé d'observer de plus près l'évolution de l'épidémie ; d'autre part, la possibilité d'instituer certains contrôles sanitaires aux frontières, ainsi qu'entre l'Hexagone et les outre-mer. c'est évidemment peu. Mais il n'en reste pas moins que l'exécutif demandait à conserver jusqu'à début 2023 un pouvoir de contrôle de certains déplacements.

Dans sa démarche habituelle de responsabilité et d'exigence, la commission des lois de notre assemblée s'est saisie du projet de loi et, suivant son rapporteur, a proposé de le remanier très substantiellement. Le texte qui en résulte opère une réelle conciliation entre la prudence indispensable face à une situation sanitaire demeurant quelque peu incertaine et l'encadrement toujours plus strict du recours par l'exécutif telle attitude a présidé au rétablissement de l'article 2, relatif au contrôle sanitaire pour les personnes entrant sur le territoire national. Ce rétablissement est le fruit d'un travail considérable de notre rapporteur, qui a construit un dispositif juridiquement robuste, très ciblé dans son application et exigeant à l'égard de l'exécutif. Il l'a fait en prenant en compte les travaux des députés, ainsi que les remarques de nos collègues sénateurs, par exemple sur la question des contrôles concernant les outre-mer. Oui ! D'autres positions historiques du Sénat s'y retrouvent également. Je pense par exemple à la consultation obligatoire du Parlement par le Gouvernement si ce dernier souhaite prolonger l'application des mesures Les travaux de la commission comprennent d'autres apports intéressants. Ainsi, le premier article du texte qu'elle a élaboré mettra un terme à l'ambiguïté que j'évoquais plus tôt en abrogeant explicitement les différents régimes sanitaires dérogatoires. Cela aurait pu aller sans l'écrire, mais c'est plus compréhensible pour tout un chacun en le gravant dans le marbre de la loi, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. L'article 2 répondra à certaines préoccupations concernant la situation des soignants suspendus. Enfin, l'article 1, relatif aux systèmes d'information contre la covid, a été complété complété par notre rapporteur avec une disposition facilitant les déplacements des Français au sein des pays de l'Union européenne. Cela se fera en prolongeant une partie du système d'information sans déroger au droit au secret médical ni effectuer de. Exactement

et permet d'éviter les formes graves d'infection, je pense que le schéma vaccinal ne constitue pas une certitude de non-contagiosité, contrairement à un test négatif fait à un instant Notre rapporteur a compris les inquiétudes des Français, qui en ont assez des différentes mesures prises depuis plus de deux ans, dont certaines furent très contraignantes ou attentatoires aux libertés, et d'autres ont constitué des obligations ne voulant pas dire leur nom. Il a toutefois pris le soin de veiller à leur protection sanitaire aux frontières et dans les territoires ultramarins et de préserver leur liberté de voyager en Europe et dans certains autres pays du monde. Il résulte de ces multiples apports un projet de loi profondément rééquilibré, et non corédigé, à même d'accompagner la sortie réelle des régimes d'exception de ces dernières années en posant de forts verrous à l'action du Gouvernement. Il faut conclure. C'est donc sans état d'âme que je voterai ce texte, comme la majorité du groupe Les Républicains.

Il y a la technique- elle a été rappelée -, il y a la politique, et il y a une réalité qui est face à nous depuis 855 jours. le ministre, nous faisons le constat d'une impuissance, d'une impréparation, d'une absence d'une politique de prévention et d'une totale incapacité à gérer une telle situation.

vous le savez mieux que nous, il y a eu quelques jours au printemps 2020 où nous avons compté les ampoules de curare, et le Doliprane est toujours sous quota Il y a eu aussi une communication totalement dépassée. On a plus parlé des « oubliés du Ségur » que des progrès réalisés dans ce cadre. Il y a eu des protocoles totalement inadaptés. En tant qu'officinal, j'ai eu l'impression de faire de la maltraitance au mois de janvier quand il fallait tester les enfants du lundi soir au vendredi matin, sans oublier le rappel ... Je vous assure qu'il y a eu une totale inadaptation face à la réalité de ce qu'on a appelé la « cinquième vague ». Tout cela a constitué la France de la défaillance. À côté de la France de la défaillance, il y a eu la France de la défiance. Il a fallu convaincre pour vacciner, alors que la France, pays de Pasteur, de Calmette et Guérin, a été dans l'incapacité de préparer un vaccin. Heureusement, après cette France de la défaillance et cette France de la défiance, il y a eu aussi la France de la résistance ! Heureusement, quelques premières lignes ont tenu les maires, les préfets, les professionnels de santé sur le terrain, le maillage officinal, le personnel des Ehpad ... Et les pompiers ; je profite de l'occasion pour le dire : oui, dans la situation exceptionnelle que nous connaissons, il faut réintégrer tous les pompiers, car nous en avons besoin La pandémie a révélé, monsieur le ministre, la fragilité de notre système de santé.

Ce qui nous a donné envie d'être professionnels de santé voilà quarante ans, c'était cet engagement, cette abnégation, ce qu'on avait dans les tripes : servir d'abord la santé, ne pas avoir une santé comptable

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de vos remarques et de la sérénité du débat, qui permet d'entendre les arguments de chacun. Vous l'avez compris, aujourd'hui, ma principale préoccupation reste la protection de nos concitoyens face à cette pandémie, qui- vous l'avez tous dit -perdure.

J'avais déposé un amendement en ce sens, car une ambiguïté demeurait. À l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle avait refusé une telle suppression, malgré la demande du député Les Républicains Philippe Gosselin. Gosselin. Les régimes d'exception, censés être temporaires, ont perduré plus de deux ans ! Alors que nous revenons dans un régime de droit commun, il est impératif de supprimer définitivement du code de la santé publique ces

article à un nettoyage législatif bienvenu, qui nous permettra d'y voir plus clair et de lever toutes les ambiguïtés, en précisant que l'ensemble des régimes d'exception que nous avons votés ces derniers mois vont bien s'éteindre d'ici quelques jours. Je profite de mon intervention

de juin dernier, l'Assemblée nationale est redevenue une véritable assemblée parlementaire, ce dont je me réjouis. En commission, elle a décidé de limiter la prolongation des régimes d'exception de lutte contre la covid-19 au 31 janvier 2023. Nous avons gagné deux mois par rapport au texte initial du Gouvernement. Mes chers collègues, je suis partagé sur cet article. En tant que médecin, je comprends la nécessité de disposer de données épidémiologiques, y compris pour vérifier la pertinence de la politique sanitaire

On sait ce qu'il faut faire pour la traiter, même si les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux, ce qui pour nous, les parlementaires, représente une certaine difficulté ! Ma conviction est que nous avons besoin d'une tout autre politique sanitaire.

Occupons-nous de ces dernières, laissons tomber cette gestion de masse, remettons le médecin au coeur du dispositif, et je pense que tout le monde s'en portera très bien ! On voit l'état dans lequel se trouve notre pays, avec les dommages collatéraux de sa gestion de la covid-19. Sortons enfin, pas uniquement dans les mots, mais dans les faits, d'une telle gestion ! Revenons à quelque chose de beaucoup plus logique, même si

Le taux d'incidence était de 3 848, alors même qu'à cette époque, on nous annonçait une couverture vaccinale de 80 % de la population, que le passe sanitaire, puis vaccinal, était en vigueur, et que le port du masque était toujours de rigueur. Alors que nous avons repris une vie normale et choisi, à juste titre, de vivre avec ce virus, nous voilà amenés, une nouvelle fois, à maintenir ou reconduire des dispositifs qui n'ont pas démontré leur efficacité, qui se sont montrés très coûteux, lourds d'un point de vue administratif, clivants d'un point de vue social et qui, selon les propres mots de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, ne sont qu'un leurre et ne protègent pas. Il faut véritablement en finir avec ce contrôle de la circulation virale. Les indicateurs de contagion ne sont plus pertinents : être contaminé n'est pas grave en soi. Le suivi centralisé de l'épidémie ne sert qu'à alimenter une épidémie de cas, et non pas de malades. Cette accoutumance du pouvoir aux moyens de traçage doit véritablement cesser.

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'oppose à la prorogation jusqu'au 30 juin 2023 des systèmes de suivi d'information et de traçage SI-DEP et Contact Covid. La loi du 11 mai 2020 avait créé temporairement ces deux fichiers nationaux pour conserver, pour une durée de plusieurs mois, les données de santé des Français qui se soumettent aux tests de dépistage du covid-19. Ces données de santé peuvent être consultées par un trop grand nombre d'acteurs, notamment par les enquêteurs sanitaires et par certains agents des services préfectoraux. Au regard des protections constitutionnelles et conventionnelles du droit au respect à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les auteurs de cet amendement alertent sur les risques de pérennisation de tels dispositifs de collecte de masse des données médicales, qui sont récoltées depuis plus de deux ans déjà, sous une forme pseudonymisée et non anonymisée. Par conséquent, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires refuse une telle prorogation, en l'absence d'études prouvant que les deux systèmes de traçage ont eu un effet réel dans sur la stratégie sanitaire de lutte contre la covid-19.

Cet amendement vise à supprimer l'article 1, qui prolonge jusqu'au 30 juin 2023 le système SI-DEP. Si l'article prévoit le consentement des personnes concernées, il s'agit d'un consentement tronqué, puisque le SI-DEP est maintenu comme le seul moyen d'obtenir les certificats demandés dans le cadre du certificat covid numérique. Il n'y a donc pas consentement. De plus, ce système n'est pas adapté à la réalité de l'épidémie et donne une vision erronée depuis l'arrivée du variant omicron, fin 2021. Le fichier devait être temporaire. Or le secret médical n'est pas assez protégé, et il y a bien une collecte massive de données médicales. recense l'ensemble des tests positifs, incluant des millions de cas asymptomatiques, ce qui entretient une épidémie de cas, et non de malades.

pour permettre aux Français de voyager en se conformant aux obligations fixées par l'Union européenne ... Ce n'est pas trop tôt ! Un autre apport très intéressant de la commission est le recueil du consentement des personnes concernées pour les seules finalités de centralisation des données de tests et de délivrance d'un certificat attestant d'une absence de contamination. Cependant, malgré la très bonne intuition à l'origine de telles mesures et leur objectif louable, nous nous interrogeons sur le découpage opéré entre les différents systèmes d'information en place

Ce texte, dont la dimension technique mérite de nouveau d'être soulignée, présente tout de même un intérêt sans véritablement froisser la susceptibilité de nos compatriotes, qui, de fait, en ont assez des contraintes, mais sont plus attentifs encore à leur sécurité.

1, à mettre un terme à plusieurs systèmes d'information clés dans la lutte contre le covid-19 à compter du 1 août prochain. Face à une épidémie qui revient par vagues- on le constate aujourd'hui -et à la forte probabilité d'un rebond au cours de l'automne ou de l'hiver prochain, il est essentiel de maintenir ces systèmes d'information, qui constituent le thermomètre de l'épidémie. Ils nous permettent de suivre son évolution et de protéger les Français. SI-DEP permet en effet de réaliser un suivi quotidien et fiable de l'épidémie, mais aussi d'anticiper son évolution en termes de volume et de variants. Contact Covid et les traitements des ARS permettent de leur côté d'assurer une prise en charge rapide des personnes concernées, un suivi, et ainsi de casser les chaînes de contamination. pas que SI-DEP génère de manière sécurisée les certificats de test et de rétablissement permettant aux Français de voyager à destination de pays qui maintiennent des restrictions à l'entrée sur leur territoire. La délivrance de ces certificats est d'ailleurs une nécessité qui résulte de nos engagements européens. Les États membres de l'Union européenne doivent être à même de délivrer des certificats covid numériques EU jusqu'au 30 jusqu'au 30 juin 2023, en vertu d'un règlement de l'Union européenne modifié le 29 juin 2022. Le Conseil scientifique et le Conseil d'État ont approuvé de telles dispositions. Ils ont tous deux considéré que la prolongation de ces systèmes pour les prochains mois était nécessaire au regard des perspectives d'évolution de l'épidémie. Je rappelle que toutes les garanties prévues aujourd'hui par la loi sont reprises par ces dispositions, afin d'assurer le droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Le Conseil constitutionnel les a déjà jugées conformes à la Constitution. La CNIL, pour sa part, s'est déjà assurée à plusieurs reprises du respect des règles applicables dans le fonctionnement concret de ces systèmes. Ils font l'objet de contrôles réguliers depuis leur démarrage en juin 2020, contrôles qui demeureront aussi longtemps que ces systèmes existeront. Je me félicite des travaux constructifs menés par votre commission des lois, qui a atteint, je le crois, le juste équilibre. Elle a en effet maintenu la date du 31 janvier 2023, qui avait fait consensus à l'Assemblée nationale, pour la prolongation à périmètre constant des systèmes d'information. Elle a en outre prolongé, en cohérence avec le règlement européen, la validité de SI-DEP jusqu'au 30 juin 2023, afin de garantir aux Français la possibilité de voyager en Europe et dans le monde. Nous conserverons ce thermomètre irremplaçable de l'épidémie jusqu'à cette date, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer dans la discussion générale.

40 000 euros par mois pour l'hébergement informatique, 40 000 euros à 80 000 euros par mois pour la maintenance et le développement de l'application, 50 000 euros par mois d'appui au support utilisateur ... Quand on demande aux Français de faire des efforts,

et à assurer ainsi un contrôle effectif des systèmes d'information mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, en l'occurrence les fichiers SI-DEP et Contact Covid, ainsi que l'application TousAntiCovid.

sur le dispositif. Cet avis a d'ailleurs été suivi d'effet, puisqu'il est intervenu au moment de la discussion parlementaire. En tant que rapporteur, j'en ai tiré toutes les conséquences. La CNIL agit donc déjà à titre préventif

peut obtenir toutes les informations utiles et a déjà le pouvoir d'ordonner la suspension des traitements de données si elle estime que leur fonctionnement ne respecte pas les règles en vigueur et d'imposer- cela a été souligné -des amendes extrêmement élevées. La CNIL a mis en oeuvre une démarche de contrôle continu sans équivalent dans l'histoire de l'institution pour les systèmes d'information covid. Elle a ainsi réalisé 48 opérations de contrôle, qui n'ont révélé aucun dysfonctionnement majeur.

et d'imposer la présentation soit d'une vaccination à jour, cher collègue René-Paul Savary, soit d'un certificat de rétablissement, soit d'un test. La commission des lois a voulu faciliter la vie des Français.

sur leur téléphone portable, en bout de chaîne, d'une information saisie par le laboratoire d'analyses biologiques sur sa vaccination ou sur son statut au regard de la contamination. Pour cela,

ont bien reconnu- je les en remercie -que le texte adopté par la commission « présente un intérêt certain quant à l'objectif recherché d'assurer à tous nos compatriotes la possibilité de voyager en Europe

votre amendement vise à supprimer la possibilité de mettre en oeuvre le système d'information SI-DEP durant la période comprise entre le 31 janvier et le 30 juin 2023. Cette possibilité a été ouverte par la commission des lois, en complément de la prorogation, à périmètre constant, mais uniquement jusqu'au 31 janvier 2023, des systèmes d'information nécessaires à la gestion de l'épidémie de covid. Le point d'équilibre trouvé par la commission des lois consiste à maintenir la mise en oeuvre de ces systèmes d'information jusqu'au 31 janvier, date qui avait également fait consensus à l'Assemblée nationale, et à prolonger la validité du seul SI-DEP jusqu'au 30 juin 2023, à l'exclusion des dispositifs de. Cette Cette prolongation a un double objectif : conserver le thermomètre irremplaçable de l'épidémie ; garantir aux Français la possibilité de voyager en Europe et dans le monde, comme cela vient d'être précisé par M. le rapporteur.

Il n'y a pas d'urgence absolue, puisque nous avons jusqu'au 31 janvier. Si, d'ici là, il il est nécessaire de prendre en compte les règles européennes pour prolonger le dispositif, nous avons le temps de le faire. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait dès à présent mois supplémentaires, alors que personne ne le demande et que ce n'est pas nécessaire, y compris pour se déplacer en Europe d'ici au 31 janvier. Cette date butoir me semble claire,

clauses de revoyure à chaque fois que le Gouvernement voulait, pour un motif légitime d'ailleurs, restreindre une liberté pour lutter contre le covid. Mais, là, il s'agit d'étendre la liberté de circuler pour les Français en Europe.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui prendre la mesure des responsabilités qui sont les nôtres. Si la situation sanitaire demeure préoccupante, nous devons désormais faire preuve de pédagogie, de prévention. Mais nous devons aussi nous adapter.

Soumettre la population à un passe pour la protéger, c'est finalement lui mentir. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'une protection individuelle, et non collective. maintenir un passe, mais, politiquement, cela revient en plus à entretenir un discours délétère sur des « citoyens irresponsables qui ne sont plus des citoyens » et à poursuivre la stratégie du bouc émissaire, dirigée contre ceux qu'on a bien envie d'« emmerder » jusqu'au bout.

apparaît superflue. Pourquoi la France bâtirait-elle un cadre spécifique alors que le droit européen a instauré le certificat numérique covid, qui permet à chaque pays membre, selon sa volonté, d'enclencher des mesures sanitaires protectrices aux frontières

Je remercie la commission et son rapporteur d'avoir réintroduit cet article 2, si curieusement supprimé à l'Assemblée nationale. Je le voterai,

contenu que la protection de nos compatriotes. Je rappelle que, dès le 26 mars 2020, je publiais un communiqué par lequel je demandais que toutes les initiatives soient prises pour faire de la Guadeloupe - mais cela valait également pour la Martinique et pour la Guyane -un isolat sanitaire. Je réitérais cette proposition dans un courrier adressé au Premier ministre le 5 avril 2020, dans le but de limiter l'introduction et la propagation du virus sur l'archipel. Je dois vous dire mon étonnement d'entendre ceux-là mêmes qui, voilà deux ans, exigeaient une protection absolue de nos frontières par des règles strictes de déplacement user aujourd'hui de mots forts et grandiloquents, dont l'écho est grand outre-mer- « discrimination », « exclusion », « stigmatisation » -, pour qualifier cette possibilité de mise en place d'un passe sanitaire, passe frontières ou certificat de voyage. où moins de la moitié des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais sont vaccinés, je considère qu'il est de bonne et sage politique, et même de salubrité publique, de permettre aux pouvoirs publics d'empêcher la survenue d'une énième vague qui ne manquera pas d'être meurtrière. Quel législateur serions-nous si nous refusions de donner au Gouvernement la faculté de protéger une population indéniablement vulnérable, potentiellement confrontée à un virus mortel ? Espérons- répétons-le

Ces mesures difficilement acceptables n'ont pas toujours été acceptées ni comprises, notamment dans les outre-mer. Aujourd'hui, nous avons une vision plus claire de l'épidémie et de ses conséquences ; nous savons mieux traiter la maladie. C'est pourquoi nous ne pouvons plus nous permettre de surréagir. En cela, la nouvelle rédaction de l'article 2 que nous propose M. le rapporteur est à mon sens équilibrée. Elle préserve la possibilité de demander aux voyageurs entrant sur le territoire national un passe sanitaire pour ralentir l'import de nouveaux variants. Ce même passe pourrait être demandé pour se rendre dans un des territoires d'outre-mer, sous certaines conditions et dans ce seul but. L'objectif affiché est clairement de protéger les outre-mer sans les isoler. C'est là toute la différence par rapport aux situations antérieures. L'application de ce dispositif ne se fera qu'en cas de risque de saturation du système de santé de la collectivité concernée et qu'après consultation de l'exécutif local et des parlementaires du territoire.

Dans ces conditions, la possibilité pour le Gouvernement de rétablir un contrôle des déplacements me semble juste et proportionnée. C'est pourquoi je voterai l'article 2 dans cette rédaction, en espérant que nos collègues de l'Assemblée nationale en feront tout autant. La parole est

puisque l'objectif était à la fois de protéger la population et de gérer un système de santé sous tension et en grande souffrance. Cette entrave aux déplacements a malheureusement causé de nombreux dégâts collatéraux sur les plans familial et personnel. Il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui d'éviter qu'ils ne se répètent que cette entrave aux déplacements a peut-être ralenti la circulation du virus, mais ne l'a pas empêchée. Alors que les vagues se succèdent, nous devons tirer les leçons de la gestion passée de cette crise. S'il ne peut plus être question de bloquer la mobilité de nos compatriotes qui souhaitent rentrer chez eux, nous devons rester responsables.

contre l'arrivée de voyageurs en provenance d'un pays où viendrait d'apparaître un variant très dangereux du covid. Pour ce qui est de notre outre-mer, nous savons à quel point son système hospitalier est fragile.

la vaccination ne protège des contaminations que dans une minorité de cas. Par conséquent, il pourrait arriver qu'une personne vaccinée montant à bord d'un avion dans un pays apparu un variant très dangereux du covid soit en réalité porteuse du virus et contaminante. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu,

qu'on ne laisse que ces solutions au Gouvernement, dans un cas- j'y insiste -tout à fait exceptionnel et improbable où il faudrait se protéger contre l'émergence d'un virus très dangereux ... Je fais appel à la raison

là au service de notre pays et au service des Français. Nous devons accepter, me semble-t-il, de maintenir des précautions qui sont extrêmement utiles, même s'il peut être déplaisant de devoir produire le résultat d'un test- personne n'apprécie de voir introduire un écouvillon dans ses narines

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité d'exiger la présentation d'un passe si les circonstances l'imposent. Or l'émergence régulière de nouveaux variants de la covid-19 à l'étranger, ainsi que l'évolution actuelle de la situation sanitaire, nécessite d'habiliter le Gouvernement à prendre ces mesures de freinage si nécessaire. Le conseil scientifique a estimé que la prolongation d'un passe frontières- ou « passe variant », dénomination plus fidèle aux débats de votre commission des lois -est proportionnée aux évolutions possibles de l'épidémie et qu'il s'agit d'un élément de la stratégie commune à bâtir avec nos partenaires européens. Cette faculté expirera en janvier 2023. Par ailleurs, si ses effets diminuent progressivement avec le temps et si elle nécessite un rappel, la vaccination confère bien une immunité efficace permettant de réduire la transmissibilité du virus et le risque de contracter une forme grave

Avis favorable également, monsieur le président.

grevé notre dispositif est l'absence de reconnaissance par l'opinion publique. Nombre de problèmes auxquels nous avons dû faire face étaient dus au fait que la légitimité du conseil scientifique était mal fondée. Il est donc important de créer une instance scientifique

présenter l'amendement n° 7. Le présent amendement vise à exclure les mineurs de 18 ans du certificat sanitaire de voyage, qui les contraindrait à la présentation d'un test de dépistage. La Défenseure des droits, Mme Claire Hédon, a rappelé à de nombreuses reprises que les restrictions imposées à l'activité et à la liberté d'aller et venir sont particulièrement préjudiciables aux mineurs peuvent affecter durablement leur développement et leur état psychique. Les restrictions de liberté ne peuvent s'apprécier qu'en considération de l'âge des personnes auxquelles la loi s'applique. Alors que le Gouvernement a choisi de lever les obligations de port du masque dans les lieux clos qu'il en appelle à la responsabilité de chacun pour se protéger et protéger les autres de la pandémie qui continue de sévir, il ne nous paraît ni proportionné ni prioritaire de faire peser ces obligations sur les mineurs.

vise à tempérer le dispositif en en excluant l'ensemble des mineurs, comme nos collègues députés avaient eu la sagesse de le faire. En matière de politique de santé à destination des mineurs, les experts valorisent l'étude et la recherche d'un équilibre

ou aux dispositifs de dépistage n'est pas optimal. Dans une logique générale, la politique de lutte contre la crise du covid devrait continuer de se concentrer sur les populations cibles, celles qui risquent d'être touchées durablement et gravement par cette maladie. La parole

titre porterait-on préjudice à des enfants ou à des jeunes qui n'auraient eu leur mot à dire concernant leur vaccination ? Enfin, il s'agirait peut-être désormais de veiller davantage au bien-être psychique de notre jeunesse, qui a déjà beaucoup souffert

un amendement de suppression de l'article 2 -que, dans des cas hautement improbables et totalement exceptionnels d'apparition dans un pays donné d'un variant du covid extrêmement nocif, il s'agirait de protéger les frontières de la France et d'interdire l'accès à notre territoire à des personnes potentiellement porteuses de ce variant et contaminantes.

fait certains de nos collègues, l'amendement de suppression. Mais on ne peut à la fois dire, d'un côté, que dans cette situation improbable hautement exceptionnelle, mais très dangereuse, il faut se protéger

Or, s'ils développent moins de formes graves- c'est largement démontré -, il est désormais acquis que, tout autant que leurs aînés, les jeunes citoyens sont des vecteurs de propagation du virus. Ils peuvent tout à fait être porteurs d'un nouveau variant. Le taux d'incidence des 10-19 ans a été récemment en forte hausse : de 144 cas pour 100 000 habitants durant la semaine du 30 mai dernier, il a atteint 759 cas pour 100 000 habitants au cours de la semaine du 4 juillet.

réintroduire ou non le certificat de rétablissement et le justificatif de statut vaccinal, je précise que la vaccination est ouverte aux mineurs depuis le 15 juin 2021 et que l'Union européenne a autorisé, pour ce public, deux vaccins, l'un développé par Pfizer-BioNTech, l'autre par Moderna. En outre, les mineurs âgés de 16 ans peuvent être vaccinés à leur seule demande, ceux qui sont âgés de 12 à 16 ans avec l'accord d'un seul parent. Et les mineurs ont accès, comme tout un chacun, au certificat de rétablissement pendant plusieurs mois suivant la réalisation d'un test positif. J'ajoute que la possibilité d'exiger un passe à partir de 12 ans est un standard international et européen. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces amendements. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.